sous les réserves d’usage. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative aux services express régionaux métropolitains

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, quatre ans après la promulgation de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM), dont le rapport annexé préconisait déjà de favoriser la réalisation de ce que nous appelions à l’époque des « RER métropolitains cher Didier Mandelli –, je suis heureux de vous retrouver pour l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative aux services express régionaux métropolitains (Serm). Je me réjouis du travail réalisé collectivement et de façon transpartisane sur ce texte. du territoire de l’Assemblée nationale, Jean Marc Zulesi, que je tiens ici à saluer tant nos échanges ont été riches et fructueux, cette proposition de loi s’est vue considérablement enrichie au cours de la navette parlementaire.

mixte paritaire. En première lecture, nous avons d’abord cherché à faire des Serm un outil au service d’une plus grande équité territoriale. Dans cette perspective, nous avions estimé indispensable d’inclure de façon systématique aux projets de Serm des lignes de cars express qui permettront, de façon sans doute plus rapide et plus souple que le mode ferroviaire, de mieux relier les métropoles à leurs périphéries les plus lointaines. Cet ajout et celui, là encore systématique, des pistes cyclables ont été maintenus dans la définition même des Serm, ce qui permet d’en faire de véritables offres de services multimodaux. avons considéré qu’il était nécessaire de remettre les territoires au cœur du processus, en renforçant le rôle des collectivités territoriales dans le choix de faire intervenir la Société des grands projets (SGP) dans leurs projets de Serm.

la répartition des compétences entre la SGP, d’une part, et SNCF Réseau et sa filiale SNCF Gares & Connexions, d’autre part. Les différents stades de la navette ont contribué, je le crois, à lever un certain nombre d’ambiguïtés, tout en nous permettant de ne pas « archipéliser » le réseau ferré national, dont le gestionnaire d’infrastructures reste et restera SNCF Réseau. Enfin, nous avons enrichi le texte, pour préciser le modèle économique et financier des Serm.

Ce rendez vous a été confirmé en commission mixte paritaire, de même que la création d’une tarification spécifique pour les circulations réalisées dans le cadre des Serm. Le niveau des péages ne saurait constituer un frein au développement de nouvelles offres de transport collectif dans nos territoires. a également maintenu le principe consistant à annexer au contrat de performance entre l’État et SNCF Réseau le programme triennal des investissements du gestionnaire d’infrastructure. Si beaucoup de chemin a été parcouru depuis le dépôt de ce texte à l’Assemblée nationale, il reste encore beaucoup à faire

Gardons en tête, mes chers collègues, l’exemple quelque peu préoccupant du Grand Paris Express. Les 765 millions d’euros prévus dans le cadre des contrats de plan État région sont, certes, un premier signal encourageant, mais ils ne devraient permettre tout au plus que de financer quelques études. Nous sommes là bien loin des enveloppes nécessaires pour atteindre nos objectifs. Je place beaucoup d’espoir, monsieur le ministre, dans la conférence de financement que je viens d’évoquer ; je souhaite qu’elle apporte un certain nombre de réponses à une équation financière qui comporte encore de nombreuses inconnues. Les transports sont un secteur de temps long, ce qui suppose de fixer un cap clair et de disposer d’une certaine visibilité en matière de financement. En parallèle, je me réjouis que le projet de loi de finances pour 2024 prévoie une augmentation du plafond d’emplois de la SGP, même si ce n’est certainement pas suffisant. Je forme en tout cas le vœu que cette dynamique se prolonge dans les années à venir, tant les besoins iront croissant. Vous pouvez compter sur nous pour y veiller. Au delà des annonces au coup par coup, une nouvelle loi de programmation des infrastructures de transport doit, comme vous le savez, monsieur le ministre, constituer

Madame la présidente, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs,

par la commission mixte paritaire. Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés

secrétaire d’État chargé des transports, affirmait déjà la volonté du Gouvernement de « doter les métropoles de liaisons transversales rapides, fréquentes et interconnectées ». Aussi la présente proposition de loi vise t elle à accélérer les projets et la réalisation rapide de ces services express régionaux métropolitains. Une nouvelle fois, le Parlement vient au secours du Gouvernement pour aider à concrétiser les annonces du Président de la République… En première lecture, grâce à l’excellent travail du tout aussi excellent rapporteur Philippe Tabarot, nous avons modifié ce texte sur plusieurs points essentiels. Sans être exhaustifs, nous avons notamment rendu systématique l’inclusion d’une offre de cars express et de réseaux cyclables au profit des territoires les plus éloignés du centre des métropoles. Parallèlement au renforcement des dessertes ferroviaires, il est indispensable d’offrir aux usagers une offre multimodale de transports collectifs publics. Nous avons également renforcé le rôle des collectivités territoriales. On ne saurait trop le répéter, il n’existe pas de modèle unique que nous pourrions dupliquer : les Serm doivent être pensés à l’échelle de chacun des territoires concernés, et ils ne se développeront pas sans l’engagement fort des acteurs locaux. Ainsi que cela a été souligné à plusieurs reprises, ces derniers n’ont d’ailleurs pas attendu ce texte pour commencer de beaux projets, dont beaucoup peinent malheureusement à aboutir faute de financement.

lutter contre l’artificialisation des sols, faire en sorte que nos transitions s’inscrivent dans un aménagement du territoire écologiquement et socialement plus juste, permettre une offre de transports dans des territoires aux spécificités très différentes. le ferroviaire offre une solution extrêmement intéressante. Avant d’aller plus loin, je souhaite saluer le travail effectué par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, et particulièrement par son rapporteur. Plus largement, je salue le travail réalisé par les deux assemblées, qui sont au rendez vous des sujets structurants pour notre société. En première lecture, notre groupe avait soulevé plusieurs points, sur lesquels je souhaite revenir rapidement, car ils sont indissociables, à notre avis, du succès des Serm.

Dans cette logique structurante, il conviendra de cibler la desserte de certaines gares RER et Transilien pour assurer la connexion entre le rail et la route, qui relèvera du ressort de la SGP, de SNCF Réseau

Comme nous avons l’habitude de le répéter dans notre groupe, les acteurs de terrains sont le plus à même de régler les problèmes de terrain. Nous avons bien pris note de la volonté du Président de la République de développer ces services de mobilité de manière décentralisée, et nous souscrivons à ces objectifs.

du retour sur expérience absolument formidable accumulé par la Société du Grand Paris dans le cadre du Grand Paris Express. Peu de pays, de métropoles et même d’entreprises peuvent se prévaloir d’avoir mené de front la construction de quatre nouvelles lignes de métro et le prolongement de deux d’entre elles,

Cette évolution législative permettra à la SGP de dépasser son statut initial, d’utiliser son expérience, afin que les grandes métropoles françaises bénéficient du même savoir faire que celui dont bénéficieront bientôt – j’en suis convaincu – les Franciliens. En outre, cette évolution permettra de sécuriser les carrières des collaborateurs de la SGP, qui pourront poursuivre ce grand dessein écologique que constitue le développement de transports publics efficaces aux quatre coins de l’Hexagone. Je suis convaincu que le développement des services express métropolitains peut rapidement prendre une ampleur importante, à condition de réunir plusieurs prérequis essentiels. Au sein des groupements d’intérêt public (GIP) locaux qui piloteront le développement des Serm, le dialogue constant et le travail en bonne intelligence entre tous les acteurs seront primordiaux. Je fais confiance à la SGP et à SNCF Réseau pour mettre en commun leurs forces mutuelles et pour créer les synergies à même de déployer le plus efficacement possible des solutions de transports efficaces. En outre, le législateur a souhaité confier, à juste titre, le pilotage de ces groupements d’intérêt public aux collectivités locales, en l’occurrence aux métropoles ou aux régions. Il faudra donc, toujours en s’inspirant de l’expérience du Grand Paris, que les opérateurs publics que sont la SGP et SNCF Réseau fassent preuve d’une transparence totale et d’une fluidité absolue dans leurs échanges avec les collectivités à la tête des projets. Si nous voulons que les Serm soient un succès, comment ne pas à nouveau évoquer le sujet du financement ? Monsieur

indispensable de permettre à ces collectivités soit de percevoir des ressources déjà existantes, soit de lever en propre de nouvelles ressources. Je me réjouis par avance de l’application de l’article ajouté par la commission de l’aménagement du territoire et du

qu’il existe également un problème de financement de l’opérateur SGP. Nous avons eu vent du fait que le plafond d’emplois appliqué à la SGP en tant qu’opérateur de l’État ne serait pas ou peu relevé, alors même que le législateur élargit considérablement le cadre de ses missions. Je suis sûr, monsieur le ministre, que vous conviendrez sans peine que si ce plafond d’emplois n’était pas relevé dans la version finale du projet de loi de finances pour 2024, cela susciterait une incompréhension le Grand Paris Express sera progressivement livré, ce qui libérera des emplois. Mais, dans l’intervalle de temps qui nous sépare de ces livraisons, les études préparatoires des Serm vont avoir lieu, notamment au moyen des fonds alloués dans le cadre des contrats de plan État région. Ces études mobiliseront nécessairement la SGP, alors même que la livraison des ouvrages du Grand Paris nécessitera la plus grande attention

très vite une solution à ce problème. Une fois donc ces non minces obstacles surmontés, il sera temps pour tous les acteurs de se mettre au travail, afin d’offrir à nos grandes métropoles des réseaux de transport répondant aux meilleurs standards mondiaux. Notre pays est une grande nation de transports, et nous disposons d’acteurs absolument remarquables dans ce secteur. Je n’ai aucun doute qu’ils auront tous à cœur, comme le législateur, d’envisager ces Serm comme un grand dessein national industriel et écologique.

Cet essor puissant ne correspond pas à une volonté nouvelle, mais a déjà connu des annonces et des échecs. Dès 1995, l’idée de RER en province surgit, mais elle est vite reléguée par d’autres priorités à grande vitesse.

dernier un déploiement du réseau pour dix métropoles et que le dernier rapport du COI ne précise cette ambition au cœur de ses recommandations. Des intentions, des annonces, mais qu’en est il concrètement ? Aujourd’hui, une dizaine de projets sont identifiés,

Nos grands bassins de transport sortiront de la mobilité subie du tout voiture lorsque l’offre de TER, de transports publics et de cars express sera attractive, parce qu’elle sera continue, cadencée et bien connectée avec les mobilités durables de rabattement de premier et de dernier kilomètre que sont le vélo, le covoiturage et l’autopartage. C’est ce développement

Le texte comprend des dispositions innovantes et pertinentes pour permettre le déploiement des Serm, garantir leur maillage territorial et la multimodalité, y intégrer de façon cohérente les réseaux des différents modes de transport et

à l’interopérabilité billettique, et à condition de diffuser l’information auprès des voyageurs, l’on renforcera la fluidité à laquelle aspirent les usagers. Notre groupe est satisfait de la mention claire du caractère « gratuit » de la remise des nouvelles infrastructures à SNCF Réseau. Nous espérons que la question des péages ferroviaires sera effectivement reconsidérée,

Personne ne peut plus nier qu’il est nécessaire de construire des trajectoires financières afin d’assurer les coûts d’exploitation devant les fortes augmentations de services et les éventuels investissements nouveaux.

Sortir des énergies fossiles d’ici à 2050, voilà le chantier prioritaire. Il y a donc urgence à trouver des alternatives écologiques et économiques à la voiture et au camion. Pour cela, le transport ferroviaire est devenu la pierre angulaire de la stratégie du Gouvernement en matière de réduction des émissions.

Aujourd’hui, des moyens importants sont enfin annoncés pour faire du ferroviaire une grande cause nationale. Comme je l’avais expliqué ici même en première lecture, cette proposition de loi va dans le bon sens. Les services express régionaux métropolitains permettront de matérialiser un véritable maillage de transport dans nos grandes agglomérations. Inscrire l’intermodalité au cœur de ce projet doit également permettre à ces services de se substituer à la voiture.

du COI, pas moins de 15 milliards à 20 milliards d’euros sont nécessaires dès maintenant pour développer les lignes, investir dans l’acquisition de matériel roulant et anticiper les futures dépenses d’exploitation.

100 milliards d’euros seront investis d’ici à 2040 pour lancer une « nouvelle donne ferroviaire », mais combien seront réellement destinés au financement de services express régionaux métropolitains ? Par ailleurs, nos débats autour de ces futurs services ne doivent pas occulter la situation préoccupante des lignes du quotidien et du fret ferroviaire. Le droit à la mobilité doit être garanti partout, que l’on habite une métropole ou un territoire rural.

Le fret ferroviaire n’est pas en reste : la part du rail dans le transport de marchandises a été divisée par deux entre 2006 et 2019, au profit du transport routier, pourtant bien plus polluant. Certaines lignes essentielles pour les entreprises sont même remises en cause, faute de financement. Je pense ainsi à la ligne de Flamboin Gouaix à Montereau, en Seine et Marne : l’État demande à l’entreprise Cemex de trouver 40 millions d’euros pour pérenniser la desserte. Pourquoi sacrifier cette ligne et les emplois qui vont avec ? avec ? Le groupe CRCE K a porté ce débat sur les moyens durant l’examen du projet de loi de finances pour 2024. Il a proposé d’allouer, dès cette année, 3,9 milliards d’euros au ferroviaire : c’est la seule façon de faire vivre cette nouvelle donne que vous appelez de vos vœux.

vous avez aujourd’hui la possibilité de soutenir réellement cette alternative que nous appelons de nos vœux. Nous avons envie de vous croire ; ne décevez pas les millions de Françaises et de Français qui ont besoin dès aujourd’hui de se déplacer dans de meilleures conditions, tout en préservant notre environnement. La parole

Cette proposition de loi est bienvenue et, à l’image du groupe du RDSE, elle a su s’affranchir des clivages idéologiques et partisans au bénéfice de l’intérêt général, de la transition écologique et de l’équilibre entre nos territoires.

de l’urgence climatique et de la fracture économique, sociale et territoriale qui s’accroît entre deux France, l’une rurale, l’autre urbaine, espérons que le déploiement des services express régionaux métropolitains sera maintenant rapide et efficace.

de fractures territoriales. À propos d’inclusion, le groupe du RDSE se félicite de ce que l’accessibilité des Serm soit renforcée. En effet, grâce à un amendement de Nathalie Delattre, les gares et pôles d’échanges créés ou adaptés dans leur cadre comprendront des aménagements permettant l’accès, le déplacement et l’information des personnes en situation de handicap. au delà des inégalités territoriales que cette proposition de loi vise à gommer, il est nécessaire de réduire parallèlement les inégalités entre individus, que les personnes en situation de handicap subissent quotidiennement.

Un projet d’une telle dimension ne saurait en effet se faire sans l’avis des maires et les décisions prises ne sauraient aller à l’encontre des intérêts locaux. Il est important que le maillage territorial des futurs Serm soit réalisé selon des critères objectifs et précis. C’est pourquoi les acteurs locaux doivent avoir toute notre confiance quant à l’élaboration du périmètre le mieux adapté à leur situation. L’enjeu de ce texte excède la seule mobilité : il s’agit de construire ensemble l’aménagement durable des territoires où liberté d’action, flexibilité et souplesse opérationnelles devront être les nouveaux dogmes.

la mise en place d’une tarification spécifique des péages ferroviaires et la prise en compte des enjeux liés à la montée en puissance des zones à faibles émissions. Il s’agit de la concrétisation d’une promesse du Président de la République, avec un budget de près de 800 millions d’euros acté dans le budget 2024. Cette première enveloppe doit permettre d’amorcer les projets. À celle ci s’ajoutent les investissements très importants réalisés dans les contrats de plan État région. Pour ce qui concerne la question du financement de ces services, une conférence nationale, dont l’organisation est inscrite dans la proposition de loi, se tiendra avant le 30 juin 2024. Finalement, ce texte, qui arrive en fin de navette, organise juridiquement le déploiement des Serm dans plusieurs grandes villes en France, en accroissant la part du transport ferroviaire dans les déplacements du quotidien, avec l’impératif d’une déclinaison spécifique à chaque profil territorial. L’objectif est que chaque collectivité concernée puisse s’approprier le dispositif et l’adapter à ses caractéristiques.

La Première ministre le rappelait en février dernier, lors de la présentation du plan d’avenir pour les transports, ce sera « lorsque nos concitoyens pourront trouver un transport en commun régulier, facilement accessible et fiable qu’ils pourront réduire leur usage de la voiture. » Ce dispositif y contribuera

À quand le Paris Brest ? C’est une grosse accélération, vous l’avez dit, alors que la France vise dix lignes de nuit d’ici à 2030. Mes chers collègues, je le constate, nous sommes sur de bons rails ! Le groupe RDPI votera pour ce texte. La parole

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je suis le dernier intervenant de cette petite, mais très belle aventure législative, même si le fait de passer par une proposition

qui, grâce à son colloque du 16 octobre dernier, a grandement contribué à renforcer les liens entre députés et sénateurs, entre majorités et oppositions. Mes chers collègues, voilà un peu plus d’un an, alors que nous étions en pleine préparation budgétaire, le Président de la République annonçait par surprise

qui se tiendra dans les six mois ! Alors que l’ensemble des acteurs, à commencer par les collectivités, crient au manque de moyens, nous attendons toujours de savoir de quel côté tombera la pièce du 49.3, stress stress annuel insoutenable, alors que nous savons tous ici que le temps des mobilités est un temps long, qui souffre des à coups et des tête à queue. D’où la nécessité de disposer d’une vision claire, de compétences claires et de plans de financements clairs.

de nouveau en garde le Sénat, comme je l’ai fait le 23 octobre dernier : le danger est grand que s’accentuent les fractures sociales et territoriales avec le développement des Serm dans les seules métropoles, si l’on ne prend pas correctement en compte

une offre complète de services s’appuyant sur les logiques de rabattement depuis le vélo et la voiture individuelle « socialisée » – covoiturage, autopartage – vers les transports plus lourds

promulguée. Nous pouvons collectivement nous féliciter d’avoir œuvré à sa réussite. Son auteur, notre collègue Vincent Capo Canellas, a su tirer les conclusions législatives de la mission de préfiguration sociale confiée par Île de France Mobilités

Grâce aux auditions et à l’examen en commission, nos deux assemblées ont fait évoluer le texte pour conforter la sécurité juridique des dispositions sans toutefois en modifier l’architecture. Je sais la réticence, voire l’opposition d’une partie de l’hémicycle à se prononcer en faveur de cette je rappelle que la question posée n’est pas celle de l’approbation ou du rejet de l’ouverture à la concurrence. Ce débat est tranché depuis près de quinze ans ! Le processus est enclenché et les acteurs s’y préparent, qu’il s’agisse de la RATP, des entreprises de transport ou des salariés.

Lors de l’examen parlementaire de la LOM, le législateur a confié cette mission à l’Autorité de régulation des transports (ART). Les députés, partant du constat que les moyens humains et budgétaires du régulateur ne progressaient pas au rythme de l’élargissement de ses missions, ont supprimé dans cette proposition de loi En procédant ainsi, le règlement des différends serait revenu au juge civil ordinaire, ce qui aurait contribué au doublement, voire au triplement du délai moyen de jugement. Ce n’était tout simplement pas concevable étant donné le caractère extrêmement sensible et épineux de ces litiges. Nous avons obtenu gain de cause au terme de la CMP, mais cette victoire nous engage. Elle nous oblige à faire preuve de vigilance sur les moyens de l’ART et sur sa capacité à mener à bien l’ensemble de ses missions avec la rigueur et l’excellence que nous sommes en droit d’attendre de toute autorité administrative indépendante. Les craintes du rapporteur de l’Assemblée nationale, Bruno Millienne, sont fondées. Il nous appartiendra donc de veiller à l’adéquation des moyens de l’ART avec ses missions en vérifiant que certaines ne s’exercent pas aux dépens d’autres. Notre commission sera particulièrement attentive à ce que le nouveau président, Thierry Guimbaud, tout juste nommé dans ses fonctions, contribue à renforcer la capacité de l’Autorité de front l’ensemble de ses missions. J’en appelle également à la responsabilité du Gouvernement afin que les décrets d’application prévus dans le texte soient rapidement publiés. Puisque le législateur a examiné et adopté ce texte en à peine un trimestre, nous attendons la même célérité de l’autorité réglementaire pour rendre l’ensemble des dispositions de la loi applicables dans les meilleurs délais. Avant de conclure,

C’est l’objectif de cette proposition de loi, qui arrive en fin de navette parlementaire grâce à une commission mixte paritaire conclusive. Je salue le travail réalisé par les deux chambres du Parlement et par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat,

sportif le plus important au monde, il était fondamental d’aménager l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP sur deux points principaux : la date de sa mise en œuvre et les conditions de travail des salariés concernés.

à Sénart, à Fontainebleau, à Bussy Saint Georges, à Lagny sur Marne, dans le pays briard ou dans la communauté de communes Moret Seine et Loing, l’application des nouvelles délégations de service public issues de la procédure de mise en concurrence avait révélé de nombreux dysfonctionnements, en place avait été mal préparée et mal encadrée. Si le constat était partagé sur ces travées, les conséquences que nous en tirions étaient bien différentes selon que l’on se situe à la droite ou à la gauche de l’hémicycle.

En ce sens, l’adoption conforme de l’article 4, qui organise la possibilité d’une mise en œuvre entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2026, prouve qu’un aménagement était nécessaire. La flexibilité dans l’ouverture à la concurrence est

Nous connaissons les difficultés auxquelles la RATP est confrontée au sujet des recrutements, et notre texte peut aider – nous le souhaitons – à lever les réticences de certains candidats. À ce titre, je salue les réflexions menées à l’endroit des conditions de travail des conducteurs de bus d’Île de France, du transfert des salariés – l’enjeu est important –, des mandats des représentants du personnel de la RATP durant la transition ainsi que des remises de biens. Je me félicite que les principaux apports du Sénat aient été préservés, particulièrement en ce qui concerne les compétences de l’Autorité de régulation des transports en matière de règlement des différends.

Il comporte des avancées pour les agents de la RATP tout en contenant les précisions nécessaires à la mise en œuvre d’une ouverture à la concurrence déjà engagée. Je remercie notre rapporteur,

Prévue pour le 1 janvier 2025, l’ouverture à la concurrence constitue un défi technique, opérationnel et social d’une ampleur inédite. Pour assurer la réussite du processus, j’ai déposé ce texte en vue de garantir à la fois la continuité

est en large partie le fruit du dialogue social mené par MM. Bailly et Grosset, sur un sujet particulièrement sensible. Nombre des recommandations et des solutions qu’ils ont préconisées sont reprises pour faciliter le transfert des salariés dans le respect de l’équité concurrentielle et en assurant la meilleure qualité de service possible, le tout dans un cadre social exigeant. Je tiens à rappeler à tous que ce texte n’institue pas l’obligation de mise en concurrence, comme l’a souligné M. le ministre. Il en corrige simplement les modalités. Le débat sur l’ouverture à la concurrence a été arbitré voilà plus d’une décennie, lorsqu’un gouvernement, au demeurant de gauche, et une majorité régionale de même sensibilité ont négocié sa mise en œuvre avec la Commission européenne, après le vote de la loi du 8 décembre 2009.

de la Cour de justice de l’Union européenne. Aujourd’hui, ni la région Île de France ni la RATP n’en contestent le principe. Je le rappelle, il s’agit d’une ouverture à la concurrence, et non d’une privatisation, puisque le donneur d’ordre, Île de France Mobilités, reste une entité 100 % publique. Ce texte est animé par l’intention de faire en sorte que le processus d’ouverture à la concurrence soit équitable, socialement juste et améliore la qualité du service, dans l’intérêt des usagers du quotidien. Il s’agit de veiller à la continuité du service public, mais aussi aux conditions de transfert éventuel des salariés. Nous fluidifions le processus et prenons mieux en compte la situation des salariés, avec un aménagement du calendrier raisonnable et respectueux du cadre réglementaire européen. Ce texte vient donc sécuriser juridiquement le cadre normatif en vigueur sur l’ouverture à la concurrence. Il apportera des garanties à tous les acteurs, en particulier aux 19 000 salariés, mais aussi aux voyageurs, qui attendent le maintien de la qualité du service rendu sans risquer de voir l’ensemble du réseau basculer en une nuit, avec tous les enjeux opérationnels afférents. Je pense notamment à la notion de centre bus visant à garantir aux agents affectés à un centre bus l’absence de mobilité géographique contrainte. Nous prenons aussi en compte la situation des salariés qui verront, demain, leur mission assurée directement par IDFM, en tant qu’autorité concédante, notamment pour ce qui concerne les fonctions de supervision du réseau. Ce travail a été fait dans l’objectif de trouver les meilleurs compromis possible en concertation avec l’ensemble des acteurs. Il s’agit d’un équilibre subtil. Comme je l’ai déjà dit, nous sommes loin des discussions de principe ou de doctrine, et nous nous efforçons d’être proches des réalités.

qu’il s’agisse de la préservation des conditions de travail des salariés, de l’intérêt des usagers ou de la continuité du service public. La LOM prévoyait à l’origine ce changement pour le 1 janvier 2025. À un an de l’échéance, chacun s’accorde à le reconnaître, les conditions matérielles, économiques et sociales d’une telle transformation ne sont pas réunies. La loi de 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires laissait aux AOM la possibilité de choisir entre une ouverture à la concurrence ou une régie publique régionale. l’option de la régie publique n’a jamais été sérieusement étudiée, ce qui est bien dommage ! Ce modèle n’aurait il pas été adapté à l’ensemble multimodal interconnecté que constitue le réseau de la RATP ? En tout cas, la réglementation européenne ne l’aurait pas empêché. Mettre en concurrence des éléments de cet ensemble multimodal, c’est toucher à un équilibre déjà bien fragile, et s’assurer des problèmes de coordination, de maintenance et de continuité de service. Les syndicats tirent la sonnette d’alarme. Les quelque 19 000 agents concernés sont inquiets quant à leur transfert aux différents opérateurs.

Or nous devons garantir l’attractivité des transports publics du quotidien. Leur développement est un sujet majeur si nous voulons assurer un report modal vers les mobilités décarbonées. Le défi est donc grand pour la région Île de France, qui s’apprête à absorber d’importantes charges d’exploitation supplémentaires et à entamer la nécessaire transition énergétique d’électrification d’électrification des bus. Outre la multiplication des opérateurs, qui sera source de complexité, l’attribution des lots pour cinq ans sera source d’instabilité. du document d’allotissement dont nous ne pouvons mesurer la pertinence, puisque son contenu précis est inconnu à ce stade ? Jusqu’à la fin de 2026, tous les deux mois un lot nouveau est alloué. Il paraît difficile, à une telle cadence, de garantir à tous des conditions de transfert « équitables, justes et bénéfiques lots ou treize lots et des lignes ou dépôts « éclatés », on peut se préparer à de sacrées complications. Ces lots seront ils équilibrés et viables ? Cela n’a rien d’évident ! La compétence de l’Autorité de régulation des transports en matière de différends concernant le nombre de salariés transférés avait été supprimée à l’Assemblée nationale. Le Sénat a tenu à réintégrer l’ART comme autorité compétente. C’est fort bien, mais encore faudrait il qu’elle soit dotée de moyens à la hauteur de l’ensemble de ses missions. M. le rapporteur a raison d’insister sur cette nécessité.

Pourquoi ne pas avoir tiré les leçons de ces dysfonctionnements ? L’expérience le montre, l’ouverture à la concurrence occasionne des problèmes. Pourrons nous les surmonter en nous empressant, sitôt passés les jeux Olympiques ? Pour toutes ces raisons, notre groupe ne votera pas ce texte. La parole

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd’hui pour examiner la proposition de loi relative à l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP. Le Sénat et l’Assemblée nationale ont proposé des dizaines d’amendements à ce texte ; malheureusement, tous ont été rejetés. Je regrette que nos propositions de bon sens n’aient pas été entendues dans le cadre d’une procédure bizarrement accélérée. Dans le même temps, à quelques mois des jeux Olympiques, les Franciliens ont connu ces dernières semaines des conditions de transport déplorables. IDFM et sa présidente, Mme Valérie Pécresse, ont ainsi déploré une « nouvelle dégradation des services de transport » et ont rappelé à la RATP et à la SNCF la « nécessité de remonter la pente Tous ceux qui prennent les transports en commun en Île de France peuvent être d’accord avec ce constat. Malheureusement, la situation ne devrait pas s’arranger avec l’adoption de ce texte, et Mme Pécresse ne devra pas échapper à sa responsabilité.

Rappelons le, la RATP a été créée en 1949 pour répondre à la désorganisation totale du réseau de transports, alors géré par plusieurs entreprises privées. Cette proposition de loi nous ramène ainsi tout droit à la fin du XIX siècle. Au moins, avec ce texte, vous aurez réussi à inventer la machine à remonter le temps Le risque est donc d’accentuer encore davantage – oui, c’est possible ! – la galère dans les transports. En effet, les exemples d’échecs d’une ouverture à la concurrence sont multiples. Dans le secteur de l’énergie, plus de vingt ans après la première dérégulation, les tarifs ont augmenté en même temps que la précarité énergétique. Dans le secteur du fret ferroviaire, la part du rail dans le transport de marchandises a été divisée par deux entre 2006 et 2019, au profit des transports routiers, bien plus polluants.

Les leçons de la privatisation du réseau Optile n’ont pas été tirées. Voilà deux ans, pour remporter les appels d’offres, les sociétés de transport ont rogné sur les acquis sociaux et les conditions de rémunération.

des grèves dans plusieurs dépôts – Saint Ouen l’Aumône, Beauchamp, Argenteuil, Saint Gratien, Genainville ou Magny en Vexin – pour arracher des accords sociaux encore insatisfaisants. Aujourd’hui, ces mêmes sociétés alertent : la maquette économique n’est pas réaliste. Elles demandent à revoir les conditions de rémunération du personnel

Nous le savons déjà, cette ouverture à la concurrence entraînera moins de bus, des lignes supprimées et une colère encore plus forte de la part des usagers des transports en commun, tant le réseau de bus est primordial pour garantir le droit à la mobilité et limiter le nombre de voitures sur nos routes. Encore une fois, les maires de nos communes devront faire le service après vente, seuls et abandonnés. Mais nous avons l’habitude ! Et quel destin pour les salariés de la RATP ?

Enfin, telle que rédigée actuellement, votre proposition de loi n’apporte pas de réponse à la suppression de la double garantie d’emploi et de retraite, pour les agents statutaires de la RATP. La perte de ces garanties issues de la loi LOM serait préjudiciable pour la suite de la carrière des salariés concernés.

Comme toujours, on nationalisera les pertes et on privatisera les profits ! Toute cette opération est financièrement très approximative et bien mal préparée. Pour preuve, la région a décidé d’étaler l’ouverture à la concurrence entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2026. Personne n’est dupe d’une telle manœuvre : il s’agit de reporter une contestation sociale d’ampleur après les jeux Olympiques. Avec les sénateurs du groupe CRCE K, nous pensons qu’une autre voie est possible. Nous déposerons prochainement une proposition de loi visant à reporter l’ouverture à la concurrence, faciliter la création d’une régie régionale et recentrer les activités de la RATP. Nous voterons donc contre cette proposition de loi.

créant ainsi un quasi monopole peu propice à l’innovation et à l’amélioration continue des services. L’ouverture à la concurrence des services de bus francilien est un processus initié par le droit européen et anticipé par le législateur français depuis plus de quinze Mais ces dernières années ont été marquées par des événements qui nous ont contraints à réviser le cadre légal et le calendrier établi au début du projet. L’ouverture à la concurrence d’un monopole historique d’État est un sujet qui suscite toujours de nombreux débats. Certains y voient une opportunité de modernisation, d’innovation et d’amélioration du service public, d’autres une menace pour les acquis sociaux des salariés, sans compter les inquiétudes légitimes des usagers, qui redoutent la dégradation de l’offre de service. Nous avons donc été confrontés à un défi technique, opérationnel et social d’une ampleur inédite. Il s’agissait de garantir la continuité du service public des transports, tout en permettant à de nouveaux acteurs d’entrer sur le marché dans les meilleures conditions possible. Cela a nécessité une approche prudente, réfléchie et progressive. Le travail de nos deux assemblées, réunies en commission mixte paritaire, a permis d’améliorer le texte, dans l’intérêt des voyageurs, des salariés et du service. Face à des agents de la RATP inquiets quant à l’avenir de leurs conditions de travail et des usagers attentifs au devenir d’un service public essentiel dans leur quotidien, il fallait relever le défi de proposer un texte pragmatique tenant compte des intérêts de chacun. J’avais, pour ma part, proposé un amendement visant à faire en sorte que les salariés de la RATP concernés par le changement d’exploitant ne perdent pas l’accès à leur plan d’épargne entreprise. Cet amendement, bien qu’attendu par les agents de la RATP, n’a malheureusement pas été retenu par notre assemblée. L’une des principales décisions prises dans le cadre de l’examen du texte a été l’échelonnement du processus d’ouverture à la concurrence. Cette décision, loin d’être une fuite en avant, est au contraire un gage de réalisme et de responsabilité. Elle permettra de prendre le temps nécessaire pour accompagner les salariés de la RATP dans cette transition, pour garantir la continuité du service public et pour permettre à de nouveaux acteurs de se préparer à entrer sur le marché. cet échelonnement ne suffit pas. La commission a également veillé à ce que l’ouverture à la concurrence ne se traduise pas par une dégradation de la qualité du service public. Les usagers du réseau de bus francilien ont le droit de bénéficier d’un service de qualité, quel que soit l’opérateur chargé de leur ligne de bus.

le texte d’initiative sénatoriale qui nous est présenté ce soir est le fruit d’un compromis intervenu en commission mixte paritaire voilà dix jours. Je veux ici remercier les membres de cette CMP, qui se sont réunis le 7 décembre dernier pour parvenir à cet accord attendu.

Il s’agit, dans des délais contraints – mais le cadre initial l’imposait –, d’aménager et de reporter le calendrier d’ouverture à la concurrence du réseau des autobus et autocars franciliens de la RATP.

Avec les jeux Olympiques et Paralympiques, qui se tiendront l’été prochain, le risque de désorganisation et de rupture de continuité du service était réel. Nos deux assemblées ont donc eu la volonté commune d’aboutir à un texte pragmatique, alors même que, dès le début, les convergences Accord déjà sur le report d’une échéance trop rapprochée, avec un échelonnement sur deux ans du calendrier d’ouverture à la concurrence. Accord ensuite sur la volonté d’offrir aux agents de la RATP les garanties sociales nécessaires pour répondre aux inquiétudes exprimées. Accord aussi sur la volonté d’un renforcement de la qualité du service rendu aux usagers. Les articles 4 et 8 ont été adoptés conformes, la discussion en CMP ayant porté sur six articles. Les points de désaccord qui subsistaient étaient minimes. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale aux articles 5 et 6 ont été retenus. Par ailleurs, des modifications de nature rédactionnelle, sémantique et d’harmonisation légistique ont par ailleurs été intégrées. En définitive, il ne subsistait qu’un seul point de désaccord : les modalités de règlement des différends éventuels liés au nombre de salariés transférés entre IDFM et la RATP. La LOM avait confié cette mission arbitrale à l’Autorité de régulation des transports. Pour le Sénat, il était important que l’ART continue de régler ces problématiques. Un point d’équilibre a été trouvé en maintenant la prérogative de l’autorité publique indépendante, mais en faisant courir le délai à compter de la saisine complète et en prévoyant qu’il puisse être étendu, sur décision motivée, de trois mois supplémentaires. C’est par conséquent, sur ce point comme sur l’ensemble du texte, une solution pragmatique que nous nous apprêtons à voter, synthèse entre garanties sociales, équité concurrentielle et respect de nos engagements supranationaux. En adoptant ces conclusions, nous exprimons notre volonté que l’ouverture à la concurrence se fasse dans de bonnes conditions. La parole

cette proposition de loi d’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP n’est pas un texte anodin ; nous avons eu les uns et les autres, au cours du débat parlementaire, l’occasion de le souligner.

postérieure à 2028. Nous ne sommes pas opposés par principe aux délégations de service public. Dans le cadre des collectivités où nous siégeons, il nous arrive d’en voter ; encore faut il que les conditions de réussite soient réunies.

démontrent que ces interrogations et ces inquiétudes sont parfaitement justifiées ; les organisations syndicales ont d’ailleurs rappelé aussi leur très forte préoccupation et leurs désaccords nombreux.

alors que la plus attendue des commissions mixtes paritaires tient actuellement sa réunion à quelques minutes d’ici, il nous revient de rendre compte de l’une de ses « petites sœurs » du jour,

et résilience, mais elle n’est pas pour autant secondaire. En plus de laisser la possibilité à Île de France Mobilités de reporter l’ouverture à la concurrence des bus du 31 décembre 2024 au 31 décembre 2026, cette proposition de loi déposée par notre collègue Vincent Capo Canellas apporte des solutions concrètes aux obstructions opérationnelles rencontrées dans le cadre du processus d’ouverture à la concurrence, tout en confortant les garanties sociales des personnels transférés aux nouveaux opérateurs.

régionalisée, placée sous l’autorité d’Île de France Mobilités. Ce que l’on n’explique pas assez à nos concitoyens, c’est que la concurrence peut être une émulation, une école d’humilité. Ce que l’on n’explique pas assez à nos concitoyens, c’est que le challenge fait grandir, car il est spontanément généreux. Il l’est pour les usagers, qui connaîtront, à n’en pas douter, un accroissement de la qualité de l’offre ; pour les nouveaux entrants, qui pourront développer leurs services ; pour les opérateurs historiques, qui bénéficieront du développement du marché.

du scrutin. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, c’est avec une profonde émotion que j’interviens ce soir, alors que le Sénat s’apprête à adopter définitivement la proposition de loi que j’ai déposée mois d’avril dernier avec Max Brisson, Pierre Ouzoulias et plusieurs de nos collègues de la commission de la culture, avec le soutien du président Laurent Lafon ; je les remercie tous très sincèrement. Je me félicite, sur le plan symbolique,

Vous savez à quel point j’ai fait mienne cette question de la restitution de restes humains depuis l’affaire de la tête maorie du muséum de Rouen, voilà quinze ans. Ce sujet, qui touche au respect de la dignité de la personne humaine, à l’égale

empreint d’humanisme et d’universalisme. Gardons à l’esprit les demandes sincères formulées par des communautés étrangères en vue d’honorer la mémoire de leurs ancêtres selon leurs rites et leurs traditions. Nous ne saurions les rejeter systématiquement ou leur imposer des délais exorbitants, alors que l’expérience des têtes maories a démontré que les restitutions sont l’occasion de bâtir des relations plus solides et plus apaisées et de développer de nouvelles coopérations en se penchant ensemble sur notre histoire commune.

Enfin, ce cadre apporte la garantie que les demandes de restitution de restes humains seront, à l’avenir, examinées de manière transparente et selon des critères objectifs, de manière à mettre un terme aux pratiques qui pourraient s’apparenter au fait du prince. Ce texte ne répond pas à une impulsion du moment il est le fruit d’une mûre réflexion, alimentée à la fois par le travail conduit sous l’impulsion du législateur par feu la Commission scientifique nationale des collections (CSNC) et par les travaux de contrôle que notre commission a engagés depuis 2019 sur la question C’est grâce à ce long processus collectif de gestation que nous sommes aujourd’hui parvenus à un texte équilibré, rendant possible la restitution de certains restes humains identifiés, tout en l’encadrant de manière suffisamment stricte pour ne pas remettre en cause le principe d’inaliénabilité, essentiel à la préservation de nos collections. Le texte circonscrit précisément les conditions dans lesquelles des dérogations à ce principe peuvent être accordées. C’est pourquoi la commission mixte paritaire est d’ailleurs revenue sur la possibilité qu’avaient introduite les députés de restitutions à des fins mémorielles. L’imprécision de ce terme aurait pu ouvrir la voie à une infinité de possibilités d’usages des restes humains restitués, au risque de faire perdre toute portée au principe d’inaliénabilité. Je sais, madame la ministre, que vous vous êtes engagée à préciser les contours du terme « funéraires » dans le décret d’application l’expérience acquise avec la restitution des têtes maories prouve qu’il recouvre un sens plus large que la simple inhumation ou crémation et qu’il recouvre toutes sortes de rites permettant d’honorer la mémoire du défunt, y compris la création d’un mémorial. Le texte met par ailleurs Le texte met par ailleurs en place une procédure objective et transparente apportant de solides garanties sur le caractère scientifique, juridique et impartial de l’examen qui sera fait des demandes de restitution : un comité scientifique bilatéral sera chargé d’identifier les restes humains cas de doute et le Conseil d’État aura pour mission de contrôler la décision de restitution avant son adoption. Les propositions de rédaction que j’ai introduites en commission mon homologue rapporteur de l’Assemblée nationale ont permis d’accroître l’information du Parlement dès le dépôt de la demande de restitution, et ce tout au long de la procédure, afin qu’il puisse, si besoin, lancer des travaux de contrôle approfondis. Compte tenu du caractère interétatique de la procédure mise en place, il n’a pas été possible de la transposer aux cas des restes humains ultramarins. C’est pourtant un enjeu majeur, pour lequel il est urgent que nous trouvions une solution, comme en témoigne le cas des restes humains kaliña conservés dans les collections du musée de l’Homme ; l’association Moliko Alet+Po, dont je salue la présence en tribune, en demande la restitution. L’article 2 vise à confier au Gouvernement le soin de remettre, d’ici à un an, un rapport au Parlement identifiant une solution pertinente, globale et pérenne. Madame la ministre, vous avez proposé, avec le ministre des outre mer, d’associer les délégations aux outre mer des deux assemblées à cette réflexion à laquelle il faudrait ajouter, à mon à mon sens, les commissions des lois et de la culture. L’important est que nous nous mettions tous rapidement autour de la table. Malgré son caractère consensuel, l’examen de cette proposition de loi a été complexifié par l’imminence de la troisième loi cadre, relative aux biens culturels. Je veux croire, madame la ministre, que nos discussions auront permis de mettre en lumière certaines des lignes directrices voulues par le législateur : la nécessité de dérogations au principe d’inaliénabilité limitées et parfaitement justifiées l’importance d’une procédure garantissant non seulement une expertise scientifique croisée, mais aussi un avis indépendant permettant d’éclairer l’autorité décisionnaire quant à l’équilibre à trouver entre les différents intérêts en jeu enfin, le besoin d’y associer le Parlement. D’ici là, il me paraît primordial de disposer d’un état des lieux précis et de donner un coup d’accélérateur à la politique en matière de recherche de provenance, afin que ces lois cadres puissent effectivement

Madame la présidente, monsieur le président de la commission de la culture, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, j’aimerais commencer par évoquer le chant VI de de Virgile, ce passage où son héros, Énée, descend aux enfers pour dialoguer avec son père Anchise. C’est le moment crucial, celui où le destin d’Énée se noue. Arrivé au bord du Styx, il trouve sur la rive du fleuve qui sépare les morts des vivants, une foule importante. Étonné et ému par ce tumulte, il demande à sa guide, la Sybille de Cumes : « Dis moi, vierge, que signifie ce rassemblement près du fleuve ? Que veulent ces âmes ? » La prêtresse lui répond Tous ceux ci que tu vois, c’est la foule misérable des morts sans sépulture ; […] « Et ils ne peuvent traverser ces rives effrayantes et ces flots grondants « Avant que leurs ossements n’aient trouvé le repos dans une tombe. Au cœur de ce grand poème, qui fonde le monde latin, se trouve donc la question sur laquelle vous, sénateurs et sénatrices, vous êtes penchés depuis si longtemps. C’est une question qui nous lie à ce que nous avons de commun avec l’Humanité tout entière. Ce 18 décembre 2023, la proposition de loi relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques va, je l’espère, être définitivement votée. C’est un moment historique, attendu par plusieurs peuples étrangers, par le personnel scientifique de nos institutions culturelles, par de nombreux parlementaires et, plus largement, par nos concitoyens. Le Sénat fait figure de pionnier. Dès 2002, il répond à la demande de l’Afrique du Sud en rédigeant une première proposition de loi. Le corps de Sawtche, plus connue sous le nom de Saartjie Baartman, est rendu à sa terre d’origine. En 2010, vous votiez la loi permettant la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle Zélande, sur l’initiative de la sénatrice Catherine Morin Desailly. Le changement des mentalités, tant scientifique que politique, s’est accéléré dès cette date. Un groupe pluridisciplinaire créé par le ministère de la culture et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a mené à la publication en 2019 d’un vade mecum pour la gestion des restes humains dans les collections publiques.

Ce travail de fond, long de plus de dix ans, a donc permis la convergence du travail législatif et des demandes des professionnels du patrimoine. Le temps d’une loi cadre était venu. Elle est née d’un travail transpartisan qui a mené à un texte d’équilibre entre la garantie du principe d’inaliénabilité et la gestion éthique des collections publiques. Chaque mot a été pesé. Rares sont les lois qui auront nécessité de consulter autant de conservateurs, de chercheurs, de représentants étrangers ! Je salue tout particulièrement l’engagement de la sénatrice Catherine Morin Desailly à qui nous devons tant. Sa détermination, son dévouement à cette cause, son travail en profondeur font honneur à la France. Exact ! Je tiens aussi à saluer l’implication du député Christophe Marion, qui a permis de parvenir aujourd’hui à un texte équilibré, grâce à un travail de dentelle et de précision. Le respect de la dignité humaine anime cette loi. Son écriture a été guidée par la connaissance approfondie de différentes situations relatives aux restes humains. La France regarde son histoire en face, entend les demandes des autres peuples et souhaite instaurer avec eux une nouvelle ère, ouvrir de nouveaux échanges culturels en ayant contribué à apaiser les mémoires douloureuses. Les commissions bilatérales sauront étudier avec rigueur et méthode l’histoire propre à chaque cas de restes humains. De cette expertise à plusieurs voix, tant historiques, ethnologiques, qu’autochtones ou juridiques, naîtra un consensus. Celui ci pourra être le fondement pour non seulement des restitutions, mais aussi des coopérations scientifiques. Les amendements adoptés par le Sénat et les modifications opérées par la commission mixte paritaire ont réaffirmé la place centrale du rapport scientifique rédigé par la commission bilatérale et ont renforcé les modalités d’association du Parlement à ces travaux. Cet écrit concourt à assurer le respect du principe d’inaliénabilité, à garantir la qualité scientifique des démarches, mais aussi à joindre la représentation nationale au processus de restitution. C’est une base prometteuse pour l’avenir, et je vous en remercie très sincèrement. Restituer les restes humains originaires des territoires ultramarins ne pouvait pas avoir sa place dans un texte visant à cadrer les demandes de restitution d’États étrangers. Mais ce travail sera notre priorité des prochains mois. J’ai en effet annoncé que le Gouvernement lancera début 2024 une mission parlementaire sur le sujet. En lien avec la délégation aux outre mer de l’Assemblée nationale et la délégation sénatoriale aux outre mer, il aura notamment pour objectif d’évaluer le corpus des restes ultramarins conservés dans les collections publiques, de consulter les autorités administratives, politiques et coutumières des outre mer, puis d’identifier le véhicule législatif le plus approprié. Le Gouvernement tiendra son engagement : d’ici à un an, et je l’espère même avant, nous aurons, avec le ministre Philippe Vigier et les territoires concernés, identifié des solutions pour déroger à l’inaliénabilité des restes humains originaires des territoires ultramarins et pour pouvoir les restituer. Permettez moi, pour conclure, de revenir à Virgile avec le chant XI, qui suit les premiers affrontements entre les armées d’Énée et les peuples latins. Des ambassadeurs viennent lui demander la faveur de reprendre les corps des vaincus, afin qu’ils puissent être ensevelis

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous souhaitons remercier les rapporteurs, la commission de la culture et l’ensemble des parlementaires qui ont participé à l’élaboration de ce texte commun sur un sujet très sensible. Les restes humains ne sont pas des biens culturels comme les autres. Je salue l’engagement de longue date de Catherine Morin Desailly, accompagnée de Max Brisson et de Pierre Ouzoulias. Après son passage au Sénat en juin dernier, cette proposition de loi a été adoptée à l’Assemblée nationale. Elle s’ajoute aux différents textes dédiés aux restitutions. Je pense, notamment, au projet de loi visant à faciliter les restitutions d’œuvres d’art spoliées par les nazis aux familles juives. Ce sont des textes importants, qui nous honorent en tant que parlementaires et nous touchent dans notre humanité. En matière de restitution, le droit évolue progressivement ; il est l’écho des évolutions de la société, ainsi que de notre rapport à la mort et au passé. Que faire des restes humains ? C’est une question aux enjeux diplomatiques, historiques et patrimoniaux majeurs. Cela représente aussi un enjeu en matière, d’éthique, de sacré et de respect de la dépouille de nos ancêtres. Qu’il s’agisse de crânes de combattants hérités de notre passé colonial ou encore de squelettes intégrés à nos collections publiques, nous défendons le principe de la dignité humaine. Avant ce texte, les demandes de restitution étaient traitées au cas par cas. Il était temps de prévoir une loi cadre à la hauteur des nombreux défis auxquels nous faisons face, un texte permettant de faciliter les retours des restes humains, tout en clarifiant les conditions à remplir. La commission mixte paritaire (CMP) est parvenue à un accord au sujet des dispositions votées dans les deux chambres. Nous nous en réjouissons. Il est important que les mesures prévues par cette proposition de loi entrent en vigueur. Une question reste en suspens : celle du devenir de ces restes humains restitués. Les usages funéraires et culturels sont extrêmement divers en fonction des pays. De son côté, la France doit apporter un soutien accru à la recherche de provenance. Il s’agit d’être en mesure de proposer une solution digne et de réparer les éventuelles injustices. Enfin, nous l’avions déjà souligné lors de l’examen de ce texte, une vaste réflexion doit être menée au sujet de l’avenir de nos collections muséales. Comment les adapter aux évolutions des usages, aux nouvelles habitudes des visiteurs, aux évolutions technologiques ? Comment perpétuer la mémoire des restes humains et œuvres culturelles destinés à quitter nos musées ? Voilà les grands sujets qui devront faire l’objet d’une réflexion collective dans les années à venir. Notre politique patrimoniale a vocation à évoluer. Le groupe Les Indépendants – République et Territoires s’engagera pleinement dans les échanges sur ces questions essentielles.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission de la culture, madame la rapporteure et auteure de la proposition de loi, chère Catherine Morin Desailly, mes chers collègues, je partirai naturellement des derniers apports de la commission mixte paritaire au texte. Le plus notable est, selon nous, l’amélioration de l’information du Parlement à laquelle il procède, qu’il s’agisse de l’information des commissions de la culture des deux assemblées en cas de demande de restitutions de restes humains dont l’identification serait incertaine l’information des mêmes commissions dans un délai d’un mois à compter de la réception des demandes de restitution des restes humains appartenant au domaine public. Ce sont des points clés. Car ce dispositif de suivi vient répondre à la principale crainte exprimée depuis le début de nos travaux sur le sujet, à savoir qu’en créant une procédure de sortie du domaine public pour les restes humains appartenant aux collections publiques, le Parlement se dessaisirait trop largement de sa compétence. En renforçant de la sorte l’information de nos commissions de la culture, nous pouvons dire que nous parvenons à un équilibre d’un côté, le Parlement sera toujours impliqué dans l’évolution du périmètre des collections publiques ; de l’autre, il ne sera pas non plus mobilisé à tout bout de champ pour adopter telle ou telle loi d’espèce. Tel était, depuis le départ, l’objectif recherché. Vous le savez mes chers collègues, les centristes sont naturellement friands de ce type d’équilibre. Mais j’exprimerai aujourd’hui une satisfaction d’autant plus grande que l’on doit cet aboutissement législatif à la famille politique que j’ai l’honneur de représenter. Le groupe Union Centriste a été moteur pour bousculer les lignes sur cette question et faire avancer notre pays. Ainsi, les deux premières lois de restitution de restes humains votées en France l’ont été sur l’initiative de Nicolas About – cité par Catherine Morin Desailly – à l’origine de la loi du 6 mars 2002 relative à la restitution par la France de la dépouille mortelle de Saartjie Baartman, la fameuse « Vénus Hottentote », à l’Afrique du Sud. En 2010, Catherine Morin Desailly parvint à faire adopter la loi visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle Zélande et relative à la gestion des collections. Ces lois d’espèce ont eu une importance historique. Face à l’augmentation des demandes, elles ont pavé la voie vers l’élaboration d’une procédure générale permettant de restituer les restes humains sans mobiliser à chaque fois le Parlement. C’est bien ce que réclame notre commission de la culture depuis des années. Avec le présent texte, elle sera enfin entendue. Je ne peux que saluer sa détermination, d’autant que la proposition de loi que nous allons voter a bénéficié de l’ensemble des travaux menés sur le sujet depuis plus de dix ans pour parvenir à circonscrire la dérogation. Je pense aux travaux de la Commission scientifique nationale des collections menés à la suite de la loi de restitution des têtes maories, relayés par un groupe de travail pluridisciplinaire mis en place par le ministère de la culture et le ministère de l’enseignement supérieur. Ces derniers ont permis de définir les critères de restitution que nous nous apprêtons à faire entrer dans la loi. Le champ du texte est restreint aux seuls restes humains identifiés d’origine étrangère. La restitution ne pourra être accordée qu’à des fins funéraires. C’est une question de dignité. La procédure est claire et les critères sont précis. C’est ce qu’il fallait faire Je remercie donc très chaleureusement Catherine Morin Desailly d’avoir gardé le cap jusqu’au bout. Je félicite également Max Brisson et Pierre Ouzoulias. Vous l’aurez compris, c’est avec une très grande satisfaction que le groupe Union Centriste votera les conclusions de cette

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, dans un contexte géopolitique international très sombre, il est peu de dire que l’aboutissement aujourd’hui de cette proposition de loi est un message bienvenu d’apaisement international et de consensus parlementaire.

Sur les restitutions culturelles en général, nous sommes en train de changer d’ère. Je tiens donc aussi à remercier Mme la ministre de la culture du travail engagé autour de cette question. n’est qu’une première étape, mais c’est une première étape essentielle. Nous avons suffisamment dénoncé, ici, le fait du prince en matière de restitutions ; ce premier cadre est donc le bienvenu. Pour le traitement spécifique des demandes de restitution de restes humains adressées par des États étrangers, nous avions besoin d’un cadre clair et transparent. Le travail engagé il y a des années par Catherine Morin a permis d’avancer plus facilement sur des critères précis et objectifs pour justifier la dérogation au principe d’inaliénabilité, tout en répondant à l’exigence de dignité et en préservant l’expertise scientifique. Ce texte s’adresse en effet à tous les États qui demandent à la France la restitution d’ossements et autres éléments confectionnés à partir de restes humains, amassés dans nos collections publiques. Par là, nous montrons que nous avons entendu leurs demandes et que nous considérons que les lois funéraires de chaque société ou communauté humaine s’imposent à nos méthodes ou à nos visions du monde passées. Par là, nous disons notre détermination à respecter l’intégrité et la dignité due à chaque corps humain après la mort. C’est après tout un des fondements de notre humanité. Pourquoi exposer ce que d’autres ont volontairement enfoui ? Respecter les morts, c’est réconcilier les vivants. Nous disons ici notre volonté que les pratiques mémorielles et le respect des ancêtres s’imposent aux pratiques historiques ou scientifiques, même lorsqu’elles visent l’objectif universel d’un approfondissement des connaissances humaines. Comme Pierre Ouzoulias l’a exprimé, ce texte va permettre d’accompagner les conservateurs vers la sortie d’une forme de déni. Sans empêcher le progrès des sciences humaines, il vise à renouveler nos pratiques et à nous préserver de l’écueil de l’exotisme,

achever d’abolir l’exotisme de notre politique muséale. Enfin, cette proposition de loi répond aux aspirations de la société française, à son attachement à un plus grand respect du principe de dignité humaine, appliqué à toutes les personnes. Les collections publiques rassemblées dans nos musées sont le reflet de notre société. Le maintien de restes humains contre la volonté des peuples y est désormais impensable. L’équilibre trouvé dans ce texte va permettre de faciliter les restitutions de restes humains et, surtout, il va permettre à notre pays d’examiner rapidement les demandes. nos établissements s’engageront dans un travail en profondeur d’identification des restes potentiellement sensibles qu’ils conservent dans leurs collections. Enfin, de loi va permettre l’enrichissement des coopérations culturelles et scientifiques avec les États demandeurs, le comité scientifique mixte. Cette initiative parlementaire va donc nous faire réellement changer de cadre, en nous faisant entrer dans une nouvelle étape de notre coopération culturelle,

Le butin, selon l’usage de toujours, est porté dans le cortège. C’est ce qu’on appelle les biens culturels. […] De tels biens doivent leur existence non seulement à l’effort des grands génies qui les ont créés, mais aussi au servage anonyme de leurs contemporains. Car il n’est pas de témoignage de culture qui ne soit en même temps un témoignage de barbarie. Cette barbarie inhérente aux biens culturels affecte également le processus par lequel ils ont été transmis de main en main. Ainsi parlait Walter Benjamin dans son ouvrage posthume. C’est dans la prise de conscience humaniste du caractère barbare de l’exhibition morbide de vestiges humains spoliés à leurs populations d’origine que la présente proposition de loi trouve sa justification quasi philosophique. Je veux rappeler qu’il a fallu près de vingt ans pour que les têtes maories conservées au muséum de Rouen soient enfin restituées au musée national néo zélandais, grâce à la loi du 18 mai 2010. Citer cette loi me permet de louanger la fortitude et la ténacité de notre collègue sénatrice Catherine Morin Desailly et de rappeler que ce texte législatif était déjà, en quelque sorte, de portée générale, puisqu’il concernait toutes les têtes maories conservées dans des musées de France, y compris celles qui n’étaient pas encore connues au moment de sa rédaction. Déjà en 2012, le Parlement considérait que ses compétences en matière de domanialité publique l’autorisaient à instituer un régime dérogatoire pour satisfaire le respect d’un principe qu’il considérait comme supérieur au caractère inamovible des collections publiques. En droit, la présente proposition de loi n’est donc que l’extension à l’ensemble des restes humains des dispositions conçues en 2012 pour les seules têtes maories. Par une curieuse alliance, les groupes La France insoumise et Les Républicains de l’Assemblée nationale nous ont reproché de déposséder le Parlement de ses prérogatives au profit de l’exécutif. Je regrette qu’ils n’aient pas pris la peine de prendre connaissance plus avant des nombreux travaux que la chambre haute a consacrés au dossier de la restitution des restes humains. Par la présente proposition de loi, le Sénat a souhaité trancher un conflit juridique entre, d’une part, la nécessaire protection des collections publiques, assurée à la fois par le code général de la propriété des personnes publiques et le code du patrimoine, et, d’autre part, l’article 16 1 du code civil, qui dispose que « le corps humain est inviolable », et que « le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial », et l’article 16 1 1 du même code, qui précise que « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort À l’occasion de l’affaire des têtes maories, le juge administratif avait considéré que le régime de protection que leur conférait le code du patrimoine l’emportait sur le statut que leur attribuait le code civil. Par ce texte, nous renversons cette jurisprudence, en considérant que le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité du corps humain justifie une dérogation au caractère inaliénable des collections publiques. Ainsi, le Parlement, sans se dépourvoir de ses prérogatives en matière de domanialité publique, considère que les restes humains, par essence, ne peuvent pas constituer des objets patrimoniaux. Ce faisant, nous transposons en quelque sorte dans le droit français les dispositions de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée par l’Assemblée générale le 13 septembre 2007, qui reconnaissait « un un droit au rapatriement de leurs restes humains » et qui invitait les États à organiser leurs restitutions « par le biais de mécanismes justes, transparents et efficaces mis au point en concertation avec les peuples autochtones concernés.

Il restera aux gestionnaires des collections publiques, ainsi qu’à leurs tutelles de se mobiliser pour assurer, dans l’année à venir, le récolement complet des restes humains susceptibles de restitution et d’en informer leurs ayants droit. La parole

la CMP a été conclusive. Je me réjouis de cette issue consensuelle, à l’instant même où nous avons bien besoin de CMP conclusives de loi est une nouvelle étape de l’engagement de Catherine Morin Desailly, treize ans après le retour des têtes maories. Je salue sa persévérance, ainsi que le soutien de la commission de la culture, en attendant le troisième volet de la législation sur la migration des biens culturels. Après les biens juifs spoliés et les restes humains, ce dernier sera le fruit du travail réalisé par Max Brisson, Pierre Ouzoulias et l’incontournable Catherine Morin Desailly à la suite de la mission d’information sur le retour des biens culturels appartenant aux collections publiques. Pour en revenir à la restitution des restes humains, le contexte actuel, avec, par exemple, le conflit en Palestine, impose une lecture particulière, alors que nous sommes dans l’attente de libération d’otages et de rapatriements de corps. Nous ne pouvons considérer des restes humains, aussi sophistiqués fussent ils, comme des biens culturels banals. Quelle que soit la date du décès, la dignité humaine impose de respecter la dimension charnelle de la relation qui unit un corps à ses proches, par liens familiaux, par descendance ou par liens historiques, nationaux ou culturels.

Cette comparaison n’est pas inopportune et n’exploite pas une émotion immédiate pour argumenter sur un problème d’une autre échelle et d’une autre temporalité. La restitution de restes humains ne doit souffrir aucune condition juridique d’inaliénabilité de biens culturels. Les seules précautions relèvent de doutes sur l’identification, qu’un comité scientifique doit lever, Bien que ce texte associe le Parlement au travail de restitution, il ne donne que très peu satisfaction aux demandes ultramarines. En janvier 2022, notre assemblée avait pourtant adopté un texte ambitieux qui se préoccupait de la restitution des restes humains d’origine française.

Comment pouvons nous associer des restes humains à des œuvres d’art inaliénables ? D’ailleurs, l’inaliénabilité des biens doit, à mon sens, porter sur la dimension culturelle du bien, et non sur sa patrimonialité. C’est sa dimension culturelle qui lui donne un caractère universel ! Je me battrai toujours pour le faire reconnaître. Cette conception conforte la perception particulière des restes humains et de l’inaliénabilité de leur statut, que le temps que le temps ne saurait transformer en simples biens culturels. Au delà des conditions de restitution des restes humains, c’est la réflexion que nous menons sur les biens culturels que cette proposition de loi nous engage à prolonger,

de janvier 2023, la ministre de la culture, Rima Abdul Malak, avait annoncé l’arrivée imminente de trois lois cadres sur les restitutions, prévues dans le calendrier législatif. Deux de ces lois sont sur le point d’être adoptées avant la fin de l’année. La première, portant sur les œuvres issues de spoliations antisémites intervenues entre 1933 et 1945, est parue au n° 169 du 23 juillet 2023 La seconde, concernant la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques, devrait, je l’espère, être définitivement adoptée par le Sénat aujourd’hui. La commission mixte paritaire, consciente des enjeux et de l’impératif de progresser collectivement sur le chemin des restitutions des restes humains appartenant aux collections publiques, a joué un rôle primordial dans l’élaboration d’une proposition de loi cadre. Cette démarche s’inscrit dans une perspective transpartisane, rassemblant des membres de différentes sensibilités politiques pour construire un consensus nécessaire face à une problématique complexe. L’essence de cette proposition de loi découle du constat partagé, au sein de la commission, de la nécessité d’apporter des solutions claires et éthiques à la problématique des restes humains dans nos collections publiques. de la complexité de la conservation de ces éléments, la commission a reconnu le besoin d’un cadre législatif général qui facilite le processus de restitution, tout en respectant les principes fondamentaux comme celui de l’inaliénabilité l’inaliénabilité du domaine public. Le processus de création de cette proposition de loi a été marqué par un engagement transpartisan, témoignant d’une volonté commune de surmonter les obstacles actuels entravant les restitutions. Les sénateurs Catherine Morin Desailly, Max Brisson et Pierre Ouzoulias ont joué un rôle essentiel dans cette initiative, mettant à profit leurs compétences et leur expérience et, surtout, démontrant une détermination à traiter cette question de manière sérieuse et responsable. Je tiens tout particulièrement à saluer la sénatrice Catherine Morin Desailly pour son engagement sans faille depuis dix ans sur le sujet. L’approche de la commission s’est inscrite dans une recherche d’équilibre entre le respect du principe protecteur de l’inaliénabilité des collections et la réponse adéquate aux demandes légitimes de populations dont la sensibilité et la mémoire sont heurtées par la conservation des restes humains de leurs ancêtres. La proposition de loi cadre qui en a résulté incarne une approche méthodique, rigoureuse et raisonnée, s’appuyant sur la rigueur scientifique pour guider le processus de restitution. En intégrant un comité scientifique mixte pour vérifier l’identification des restes en cas de doute, le texte se dote d’un mécanisme de contrôle supplémentaire, renforçant la crédibilité du processus. L’accent mis sur la nécessité de transparence, à travers la transmission annuelle d’un rapport au Parlement, témoigne de la volonté de la commission de garantir un suivi démocratique et un contrôle continu sur l’application de la procédure. Cette transparence renforce la légitimité du processus, tout en permettant au Parlement de jouer pleinement son rôle dans la gestion éthique des collections publiques. En résumé, la commission mixte paritaire a agi de manière déterminée et consensuelle, pour aboutir à une proposition de loi cadre qui représente une avancée significative dans le traitement des demandes de restitution de restes humains. Cette initiative collective témoigne de la capacité du législateur à répondre de manière responsable aux défis sociétaux, combinant méthode, rigueur scientifique et respect des principes fondamentaux qui guident notre action. La dernière loi de restitution, qui, comme l’a annoncé la ministre Rima Abdul Malak, portera sur les biens culturels pillés durant la période coloniale, pourrait nous être soumise dans les premiers mois de 2024. Espérons que nous parvenions une nouvelle fois à un travail consensuel sur ce texte encore plus complexe. En adoptant ces propositions, nous affirmons notre engagement en faveur d’une gestion éthique de notre patrimoine culturel, respectant la dignité humaine et favorisant la coopération internationale.

et nous invite à faire preuve d’une profonde réflexion sur notre passé et à agir avec justice et respect. Je tiens tout d’abord, bien sûr, à saluer le travail remarquable et la pugnacité de nos collègues Catherine Morin Desailly, Max Brisson et Pierre Ouzoulias, dont l’engagement a été crucial dans l’élaboration de cette proposition de loi relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques. Il est temps de reconnaître que ces restes humains, bien loin d’être de simples objets d’exposition, sont les témoins silencieux de vies passées et de cultures riches et qu’ils portent souvent en eux le poids d’une histoire coloniale complexe. trop fréquemment été acquis dans des conditions non compatibles avec les valeurs de notre République, et leur qualification en tant que « biens », dépourvus souvent de tout intérêt scientifique, perpétue une vision dépassée du patrimoine matériel.

Jusqu’à ce jour, les rares restitutions ont été entravées par le caractère inaliénable des biens du domaine public, une barrière qui a limité la reconnaissance de la dignité inhérente à chaque individu, même après sa mort.

législatif. Face à la lourdeur et à la complexité du recours à la procédure législative, il était impératif de construire une loi cadre. C’est ce que nous faisons aujourd’hui. Cette nécessité est soulignée par les établissements concernés, au premier rang desquels les musées de notre pays, qui sont touchés par les débats de société, ne sont pas hermétiques aux

en adaptant ou en travaillant à leur législation. Il nous fallait être à l’heure et au rendez vous. La présente proposition de loi y répond, en créant un cadre clair et cohérent pour les restitutions futures, loin des décisions fragmentées et arbitraires du passé. Cette initiative va au delà de simples gestes symboliques. Elle incarne notre volonté collective de reconnaître un passé douloureux et de construire ensemble un avenir fondé sur un respect mutuel entre les peuples et les nations, notamment entre la France et ses anciennes colonies.

des zoos humains. Enfin, la démarche que nous officialisions aujourd’hui ne pourra pas réussir – j’insiste sur ce point – sans y adjoindre les moyens humains et financiers à la hauteur du travail colossal

que réparer les erreurs du passé : nous faisons honneur à notre pays, nous affirmons notre engagement envers une réconciliation des mémoires et nous construisons un avenir où le respect de la dignité humaine est au cœur de nos actions. Le groupe socialiste votera donc pour cette proposition de loi. La parole

de réfléchir avec ces collègues au cadre pérenne et méthodologique dont notre pays aura besoin demain pour répondre à d’autres demandes de restitutions en provenance de pays étrangers. Cette réflexion, nous l’avons voulue transpartisane. Cela était indispensable pour l’inscrire dans le temps long et l’éloigner autant que possible des passions que ce sujet sensible peut parfois déchaîner. Sur la question particulière des restes humains, notre séance de ce soir marque l’aboutissement des travaux conduits depuis longtemps par le Sénat. Les restes humains n’étant pas des biens ordinaires, leur restitution se justifie en vertu d’un principe qui n’est pas d’ordre patrimonial, mais qui tient au respect de la dignité des personnes.

Cependant, depuis lors, d’autres voies ont été empruntées, au mépris du Parlement. Ce fut le cas pour la restitution de crânes à l’Algérie. Aussi avons nous voulu, à l’occasion de notre mission d’information de 2020, proposer un cadre permettant d’échapper au fait du prince, qui veut que le Parlement vote des lois d’espèces, réduisant celui ci à une simple chambre d’enregistrement de décisions déjà prises, voire exécutées. Au travers de notre rapport et de la proposition de loi qui en était issue, nous avions alors réaffirmé l’importance du rôle du Parlement. qu’au delà des restes humains, et pour l’ensemble des collections publiques, une instance scientifique capable de porter une analyse objective sur l’origine des œuvres, leurs itinéraires et leurs conditions d’entrée dans les collections publiques était le seul moyen d’éviter vaines polémiques et réécritures historiques. ! sur ces points, nous avions été éconduits par le Gouvernement. Fort heureusement, madame la ministre, à votre prise de fonctions, vous avez renoué le dialogue en soutenant la construction d’un triptyque législatif sur les restitutions.

Oui, chaque année, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport présentant les demandes de restitutions adressées et le sort qui leur a été réservé. Oui, à chaque demande, le Gouvernement informera les commissions permanentes du Parlement chargées de la culture. Oui, les critères de restituabilité seront clairement définis. Il devra s’agir d’une demande portée par un État étranger datés d’une époque postérieure à 1 500 et appartenant à un groupe vivant dont la culture et les traditions restent actives, et dont les conditions de collecte portent atteinte au principe de la dignité humaine. Mes chers collègues, vous l’avez compris, le texte proposé fixe désormais une méthode et un cadre juridique clair, ce que nous demandions depuis plusieurs années. Projetons nous désormais, madame la ministre, vers la dernière partie du triptyque. Je vous le dis très clairement : notre positionnement du jour ne présage en rien de celui que nous adopterons lors de son examen. Pour répondre aux demandes de restitutions d’œuvres d’art, je crois que notre pays doit encore affiner une méthodologie consensuelle et transparente. Le débat existe : la France doit elle se doter d’un cadre pérenne suffisamment solide pour assumer la sortie de ces biens, ou en rester aux lois d’espèce ? Je suis à titre personnel persuadé de la nécessité d’un cadre méthodologique fixé par la loi,

inscrite dans un dialogue des cultures revivifié, la solution passera par l’inscription dans le XXI siècle du principe intangible d’universalisme de nos musées et du caractère exceptionnel de la dérogation au principe d’inaliénabilité de nos collections. Le Parlement devra, d’une manière ou d’une autre, en rester le garant. Madame la ministre, pour y parvenir, nous ne dérogerons pas à la ligne de conduite qui est la nôtre : l’établissement d’une méthode claire

La séance est reprise. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, au terme d’une année marquée par l’adoption au Sénat, à deux mois d’intervalle, de deux propositions de loi visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie, nous nous apprêtons à adopter définitivement la proposition de loi présentée par François Patriat

Je commencerai par la mesure phare de cette proposition de loi : la consécration, dans le code général des collectivités territoriales, de l’emploi de secrétaire de mairie comme un emploi de catégorie B au moins. La commission des lois du Sénat avait appelé une telle disposition de ses vœux dès le mois de mai dernier, sans pouvoir toutefois l’introduire elle même, du fait de l’article 40 de la Constitution. nous devons d’être cohérents : dès lors que nous mettons en avant le niveau élevé de responsabilités qui incombe aux secrétaires de mairie, ainsi que le large éventail des compétences attendues, nous devons reconnaître l’emploi de secrétaire de mairie comme un emploi de catégorie B au moins. gré, monsieur le ministre, d’avoir finalement intégré cette mesure lors de l’examen en séance à l’Assemblée nationale. Au 1 janvier 2028 s’ouvrira ainsi une nouvelle dynamique de recrutement, avec l’obligation de nommer des secrétaires de mairie à des postes relevant de la catégorie B au moins. Naturellement, je n’ignore pas que nous demandons, par là, un certain effort financier aux maires. Mais l’exigence d’un niveau élevé de compétences n’a t elle pas un prix ? Aussi suis je convaincue que les maires joueront le jeu. Par ailleurs, nous avons souhaité, en commission mixte paritaire, que la nouvelle dénomination de « secrétaire général de mairie » entre en vigueur dès la promulgation de la loi, sans attendre 2028. Ce changement d’intitulé participera d’une revalorisation symbolique, mais non moins importante de ce métier. ensuite évoquer rapidement l’article 2, qui prévoit une voie de promotion interne par la formation qualifiante pour l’accès à la catégorie B. Vous vous en souvenez, nous avions souhaité, au Sénat, réserver aux secrétaires de mairie déjà en poste cette voie de promotion interne dérogatoire. De son côté, l’Assemblée nationale a rétabli la version initiale de

Vous percevez sans difficulté le prodigieux effet d’aubaine qu’une telle disposition créerait. Pour limiter ce risque, la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire prévoit trois dispositions. Premièrement, seuls les fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d’avancement seraient éligibles, c’est à dire, les adjoints administratifs principaux. Deuxièmement, il ne suffirait pas d’avoir suivi la formation qualifiante, mais il faudrait l’avoir validée par le biais d’un examen professionnel qui permettrait de vérifier l’acquisition effective de compétences. Un décret précisera la nature de cette formation, ainsi que les modalités d’organisation de l’examen professionnel. Je précise d’emblée que l’organisation de cet examen professionnel reviendra en toute logique aux centres de gestion, qui organisent déjà l’ensemble des examens professionnels, de sorte que cette nouvelle disposition n’induira pas d’accroissement de charge pour eux. eux. Troisièmement, l’inscription sur la liste d’aptitude du cadre d’emplois de catégorie B ne vaudrait que pour la nomination à un poste de secrétaire de mairie. De plus, l’agent aurait l’obligation d’exercer ces fonctions pendant une certaine durée fixée par décret. Je souhaiterais vous faire part d’un regret : le texte ne prévoit aucune disposition qui bénéficierait tout particulièrement aux secrétaires de mairie, qui relèvent déjà depuis plusieurs années de la catégorie B. Au delà des secrétaires de mairie qui sont aujourd’hui en catégorie C et qui constituent près des deux tiers des effectifs actuels, il est essentiel de ne pas oublier les secrétaires de mairie relevant aujourd’hui de la catégorie B, qui représentent près d’un quart des effectifs. la majorité d’entre eux d’accéder à la catégorie A : la préparation d’un concours est hors de leur portée, tandis que les règles de promotion interne de droit commun sont rigides. Monsieur le ministre, je me permets de vous poser directement la question : ces agents là ne méritent ils pas également de bénéficier d’une disposition exceptionnelle favorisant leur promotion dans la catégorie supérieure,

je ne demande la requalification globale des secrétaires de mairie de catégorie B vers la catégorie A. Mais j’estime qu’il aurait été juste de donner un « coup de pouce » à ces agents, grâce à une disposition limitée dans le temps. Je regrette de ne pas avoir été comprise, et que nous soyons contraints d’en rester là Mes chers collègues, cette proposition de loi marque une première étape, que je vous invite à voter. Il reviendra ensuite au Gouvernement de travailler aux évolutions réglementaires, qu’elles soient propres aux secrétaires de mairie ou communes à l’ensemble des agents publics territoriaux. À ce propos, je veux rappeler, une nouvelle fois, la nécessité de revoir l’ensemble des grilles indiciaires de la fonction publique territoriale, dans le contexte bien connu de « tassement » des grilles. De même, la refonte générale des règles d’avancement pour l’ensemble des fonctionnaires mériterait également d’être menée à bien au plus vite. La parole est à M. le ministre.

à vous également, madame la rapporteure Di Folco, dont je connais l’exigence – je sais combien vous avez veillé à ce que ce texte serve strictement l’intérêt des secrétaires de mairie

« secrétaires généraux de mairie », que nous rencontrons, vous comme moi, régulièrement. Ils attendent beaucoup de ce texte,

Vous l’avez dit, madame la rapporteure, adopter ce texte aujourd’hui, c’est permettre : d’inscrire la fonction de secrétaire général de mairie dans le code général des collectivités territoriales

pour l’attractivité et l’efficacité de nos services publics. J’en suis absolument convaincu : c’est dans nos mairies et nos services publics de proximité que nous devons préparer l’avenir de nos services publics. Derrière chaque secrétaire général de mairie se trouve l’agent public de demain. Sous Sous cette proposition de loi perce en réalité le projet de loi que j’aurai l’honneur de vous présenter pour la fonction publique l’année prochaine. Formation qualifiante, reconnaissance de l’expérience, quotas de promotion, accélérateurs de carrière : voilà autant de sujets dont nous aurons l’occasion de débattre au premier semestre 2024. La Première ministre a confirmé

et son groupe, puis par l’initiative législative du président François Patriat et du groupe RDPI. Ce bouquet d’initiatives extrêmement positives ne peut que nous réjouir, car il est pertinent, indispensable, et urgent ; il est par ailleurs souhaité et attendu par les associations d’élus.

il n’y a pas d’avenir pour nos territoires sans avenir pour les élus, mais il n’y a pas d’avenir pour les territoires ni pour les élus sans avenir ni perspectives pour les personnels de la fonction territoriale. Le désenchantement de tant de maires découle aussi pour partie de leur dénuement face à la complexité de leurs missions, mais aussi à l’obligation d’infaillibilité juridique à laquelle ils sont soumis et qui repose trop souvent et pour beaucoup sur les épaules des secrétaires de mairie. Si les maires sont des inventeurs de possibles, ils ne peuvent rien sans leurs secrétaires de mairie, qui sont les chevilles ouvrières

afin d’éviter l’évasion vers des collectivités plus attractives, phénomène que nous connaissons aujourd’hui. Nous luttons aussi contre la solitude et la pression qui pèsent sur des secrétaires de mairie, qui sont souvent seuls dans les petites communes pour quelques jours, par la création d’un réseau qui permettra d’échanger des

je veux vous livrer ici les pensées du groupe GEST sur ce texte, en particulier celles de notre collègue Guy Benarroche, qui est retenu par une certaine CMP à l’Assemblée nationale… nationale… Les discussions ont bien eu lieu sur le texte – la première fois, à l’occasion de la proposition de loi de nos collègues du groupe communiste adoptée en avril.

Il est regrettable que l’unanimité obtenue au Sénat dès le mois d’avril n’ait pas suffi à la majorité présidentielle, qui a donc déposé un texte au titre similaire pour chercher à revendiquer une paternité sur ce sujet. La manœuvre nous semble pour le moins mesquine, le Gouvernement n’ayant pas jugé utile alors d’exprimer ses positions et de proposer ses solutions sous forme d’amendements. Nous y voyons le reflet d’une impréparation, voire d’une politique fluctuante et peu définie… Au sein du Parlement, le débat a donc eu lieu. Nous parlons aujourd’hui du compromis trouvé la semaine dernière en CMP. Que pouvons nous dire de ce texte ? Premièrement, le poste de secrétaire de mairie est l’un des rouages clés du fonctionnement de notre échelon local. Véritable outil d’interface entre les élus, d’une part, l’administration et les citoyens, d’autre part, ce poste, pourvu par des femmes en très grande majorité – à 94 % –, ne bénéficie pas d’un cadre ou d’un statut à la hauteur des missions qui lui sont dévolues.

intitulé, conditions d’accès, grille indiciaire – ne relèvent toutefois pas de la compétence du législateur. » La commission des lois « a donc préféré substituer aux dispositifs proposés l’instauration d’une formation initiale commune à l’ensemble des secrétaires de mairie, quel que soit leur statut, ainsi qu’une mesure visant à favoriser la promotion interne des agents exerçant ces fonctions. » Là encore, nous regrettons que le Gouvernement n’ait pas pris d’engagement sur le sujet, pas plus que sur le financement nécessaire pour l’intégration et l’avancement de la catégorie B vers la catégorie A de ces postes. Le choix d’étendre à l’ensemble des communes de 2 000 habitants la possibilité de recruter sous forme contractuelle pour ces emplois ne semble qu’un pansement sur une jambe de bois. Le temps des mesures ponctuelles doit prendre fin, l’absence de reconnaissance spécifique à ce poste ne peut plus durer. Par ailleurs, la contractualisation à plus grande échelle nous pose toujours problème. Comme les deux tiers de ces personnels exercent à temps partiel et que près d’un quart d’entre eux travaillent sur plusieurs communes, nous aurions préféré une réflexion sur la mutualisation de ce poste,

nous l’espérons courte – vers une réelle amélioration des conditions d’exercice, de recrutement et de pérennisation nécessaires au poste de secrétaire de mairie. Notre groupe votera donc

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’importance du rôle des maires n’est plus à démontrer, bien que leur statut demande lui aussi à être largement reconsidéré.

Nous arrivons aujourd’hui à une étape importante avec le vote, que j’espère unanime, de mesures qui permettront une juste reconnaissance pour les personnes exerçant cette profession avec dévouement.

outre, le recul des autres services publics dans nos territoires. Les secrétaires de mairie – des femmes, dans l’immense majorité des cas – doivent être polyvalentes en tout point. Elles travaillent, pour la plupart d’entre elles, dans plusieurs communes à la fois, parfois éloignées, cumulant les temps partiels. Elles doivent à la fois maîtriser le budget, l’état civil, les questions d’urbanisme, les marchés publics, rédiger arrêtés et délibérations, et j’en passe, tout en répondant aux demandes multiples et variées des habitants, la commune étant le premier, mais parfois aussi le dernier service public de proximité. Mobilisée depuis plusieurs mois sur ce sujet, j’ai constaté la lassitude qui peut gagner les secrétaires de mairie face à leur charge de travail, leur petit salaire, la difficulté de se faire remplacer ou de trouver des interlocuteurs, proches et à l’écoute, notamment au sein des services de l’État. Nous connaissons une crise de recrutement. Le nombre de personnes voulant s’engager dans ce métier ne cesse de diminuer, alors même qu’un tiers des secrétaires de mairie en poste partira à la retraite d’ici à 2030.

destinant à ce métier et formalisera le travail en réseau qu’elles demandent pour sortir de leur isolement. Cette proposition de loi ne devra cependant pas : je crois que tout le monde se rejoint sur ce point. Nous sommes parvenus à mieux mettre en lumière cette profession : cette lumière ne doit plus s’éteindre ! Il me semble indispensable – je rejoins en cela les propos de notre rapporteur Catherine Di Folco – de renforcer les possibilités de

véritablement rendre ce métier plus attractif. Le sujet des remplacements doit aussi être travaillé, même si j’ai conscience de sa complexité. Nombre de secrétaires de mairie peinent à partir en formation, ou tout simplement en congé, et à laisser la mairie porte close. Enfin,

nous arrivons au bout de la navette parlementaire pour ce texte qui fait l’unanimité sur les travées de notre hémicycle. Nous saluons les travaux de notre assemblée, depuis la proposition de loi initiale

À la base de ces travaux législatifs, n’oublions pas les agents eux mêmes, qui se sont pleinement mobilisés et parfois constitués en associations pour porter la voix des secrétaires de mairie dans bon nombre de départements comme le

Ce texte parle bien sûr à tous les élus de terrain et de terroirs qui connaissent l’importance du rôle des secrétaires de mairie pour le bon fonctionnement de notre démocratie locale. coopération intercommunale de Lot et Garonne, dans un département rural, voire hyper rural, selon l’expression de notre regretté collègue Alain Bertrand, je sais ce que nous devons à ces personnes dévouées, qui exercent un métier polyvalent, parfois aride, souvent ardu. Leur relation de confiance et de solidarité avec les élus est irremplaçable. En effet, les secrétaires de mairie sont les rouages essentiels des services publics de proximité, en première ligne de la demande citoyenne. Elles – 94 % des secrétaires sont en effet ! – assurent parfois les services de plusieurs communes, et pas que d’une seule, surtout dans les petits territoires, sans pour autant recevoir la reconnaissance institutionnelle nécessaire. de juillet dernier, sur l’initiative du centre de gestion de Lot et Garonne et de son président Christian Delbrel, nous avons réuni les 280 secrétaires de mairie de Lot et Garonne. Nous remettions alors officiellement les diplômes aux lauréates et lauréats du diplôme universitaire

est une initiative des quatre centres de gestion de Lot et Garonne, des Landes, de Gironde et de Dordogne, en partenariat avec l’université de Bordeaux et son antenne agenaise.

Ainsi, l’article 1 A consacre les fonctions de secrétaire de mairie dans le code général des collectivités territoriales. À compter du 1 janvier 2028, les nouveaux secrétaires généraux des communes de moins de 2 000 habitants devront relever d’un cadre d’emploi de catégorie B et ceux des communes de plus de 2 de catégorie A. Je pense qu’il s’agit là d’une reconnaissance importante pour nos agents. Les secrétaires de mairie de catégorie C, déjà en poste, bénéficieront de nouvelles voies de promotion interne pour un accès facilité à la catégorie B.

exercées. Mes chers collègues, le groupe RDSE soutiendra des deux mains ce texte, qui traite d’un vrai sujet de préoccupation pour nos élus locaux et qui apporte des solutions utiles pour maintenir la qualité de nos services publics. Jeune sénateur, c’est avec des visages et des expériences encore vives à l’esprit que je voterai pour ce texte, convaincu du bien fondé des positions défendues.

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame le rapporteur, mes chers collègues, auquel nous appartenons, nous pouvons tous, ce soir, saluer l’adoption imminente d’une proposition de loi d’une grande utilité pour nos communes rurales. Je souhaite exprimer ma reconnaissance envers les membres de la commission mixte paritaire qui ont travaillé dans l’esprit de de concertation transpartisane qui a prévalu tout au long de la navette parlementaire. Le métier de secrétaire de mairie, présent dans plus de 29 000 communes, est au cœur de nos collectivités. Cependant, il figure parmi les douze métiers les plus en tension dans la fonction publique territoriale en raison d’un déficit d’attractivité préoccupant. Actuellement, plus de 1 900 postes sont non pourvus et près d’un tiers des agents en activité prendront leur retraite d’ici à 2030, ce qui suscite une vive préoccupation quant à la continuité des services essentiels à l’échelon local. Les auteurs de cette proposition de loi ont eu une double volonté

Ce texte répond également aux besoins de formation exprimés par la profession, confrontée au manque de temps, à l’éloignement géographique des lieux de formation et aux difficultés à trouver un remplaçant pendant les absences. Les missions des secrétaires de mairie sont pléthoriques, englobant des domaines tels que la comptabilité, le droit, les ressources humaines, soulignant ainsi la polyvalence et la complexité de leur rôle. Les apports du texte issu de la commission mixte paritaire sont significatifs. En ce qui concerne l’attractivité du métier, le texte prévoit que, à compter du 1 janvier 2028, la fonction de secrétaire général de mairie sera accessible à partir de la catégorie B, plutôt que la catégorie C, marquant ainsi une avancée considérable. Les personnes exerçant actuellement cette fonction en catégorie C seront accompagnées dans leur passage de grade, soit par une facilitation pour celles qui relèvent des grades d’avancement dans leur cadre d’emploi respectif, soit par la validation d’un examen. Il est également souligné dans le texte qu’il ne devrait par la validation d’un examen. Il est également souligné dans le texte qu’il ne devrait y avoir aucune distinction dans la dénomination du métier entre les catégories A et B, la dénomination commune de « secrétaire général de mairie De plus, le texte prévoit un avantage spécifique d’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon pour les secrétaires généraux de mairie, reconnaissant ainsi l’expérience et le dévouement des professionnels en place. Enfin, le suivi de cette proposition de loi sera assuré par le Gouvernement, conformément à l’article 2 A, avec l’obligation de rendre un rapport évaluant les formations supérieures préparant au métier de secrétaire de mairie, répondant ainsi à une forte demande d’accompagnement à la formation exprimée par les professionnels. Le groupe RDPI soutient la démarche de son président François Patriat, à l’initiative de cette proposition de loi, démontre une fois de plus sa connaissance du terrain et des territoires, se positionne naturellement en faveur de cette proposition de loi et se tiendra aux côtés du Gouvernement et des collectivités pour contribuer activement au déploiement réussi de ce texte. Nous sommes convaincus que ces mesures contribueront non seulement à résoudre les défis actuels du métier de secrétaire général de mairie, mais aussi à renforcer l’ensemble de nos communautés rurales. La parole

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les travaux parlementaires relatifs à la situation des secrétaires de mairie que nous sommes appelés à conclure aujourd’hui, ont commencé au mois d’avril dernier. Eu égard à l’urgence concernant ce métier en tension, ils auraient mérité que nous puissions aboutir au vote d’un texte avant la fin de l’été. Ce ne fut pas le cas. Ce sujet nous a mobilisés de manière transpartisane et unanime. Ce résultat découle d’une prise de conscience partagée, à la suite des témoignages et des alertes que nous adressent depuis plusieurs années les maires et les élus municipaux. Aussi, je tiens à remercier nos collègues Céline Brulin et François Patriat, grâce auxquels ce sujet a été inscrit à l’agenda du Sénat. Je souhaite également saluer nos collègues Catherine Di Folco, Jérôme Durain et Cédric Vial, qui ont produit un rapport d’information de qualité sur les secrétaires de mairie au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, que préside notre collègue Françoise Gatel. Les sénateurs et sénatrices du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ont activement participé à ces travaux et soutiennent le texte issu de la commission mixte paritaire. Nous le faisons animés par le souci d’être utiles et de répondre aux demandes des secrétaires de mairie. Nous connaissons tous et toutes le rôle primordial que les secrétaires de mairie tiennent dans les municipalités. Juristes, urbanistes, comptables, informaticiens, les secrétaires de mairie sont des interlocuteurs essentiels pour les habitants, pour lesquels ils représentent le premier service public de proximité, d’ailleurs souvent le seul… Les secrétaires de mairie sont aussi des partenaires précieux pour les maires et leur équipe municipale. Véritables chevilles ouvrières de l’action publique, ils méritent toute la mobilisation du législateur, mais également et surtout celle de l’exécutif. malgré toute l’importance de cette profession, celle ci attire de moins en moins. Alors que notre pays compte aujourd’hui 23 000 secrétaires de mairie, 1 900 postes ne trouvent et plus de 30 % des postes actuellement occupés seront vacants d’ici à 2030 en raison des départs à la retraite. Je ne puis naturellement m’empêcher de penser à la situation de mon département, l’Indre et Loire : près de la moitié des secrétaires de mairie des communes de moins de 3 500 habitants seront partis à la retraite d’ici à quatre ou cinq ans. Les causes relevées par les secrétaires de mairie sont leurs conditions de travail, le manque de reconnaissance de leur statut, l’absence de parcours concret de formation face à la multiplicité des tâches à accomplir dans ces emplois, mais également leurs salaires, bien trop bas sans oublier le manque de perspective en matière d’évolution et de promotion. Le législateur a tenté de remédier à ces problèmes, dans la limite qui lui est imposée par l’article 40 de la Constitution. Aussi, le vote de cette proposition de loi, s’il est bienvenu, ne réglera pas l’ensemble des questions soulevées. C’est donc avec lucidité et en responsabilité que nous voterons ce texte,… Très bien ! … qui contient des mesures nouvelles et utiles. Nous y souscrivons, même si nous déplorons qu’une proposition de loi plus ambitieuse ne puisse être adoptée en raison de contraintes constitutionnelles. Ah… Aussi, monsieur le ministre, nous attendons avec impatience le projet de loi transversal et volontariste sur la fonction publique que vous nous avez annoncé depuis plusieurs mois déjà. De la même manière, si les élus municipaux sont bien disposés à prendre leur part en matière d’augmentation

nous avons pour habitude de mettre en avant le rôle vital des communes dans nos territoires, à la fois comme échelon démocratique de base et comme cadre privilégié de l’exercice de proximité de nombreuses compétences. En raison même de leur maillage territorial très fin, la plupart des communes sont petites et dotées de moyens limités. Dans ce contexte, les secrétaires de mairie assument souvent un rôle de cheville ouvrière indispensable au fonctionnement des communes de moins de 3 500 habitants. Leurs tâches vont de l’accueil du public à la gestion des opérations funéraires, à l’instruction de demandes officielles, voire à la passation de marchés publics. Principaux collaborateurs des élus municipaux, se partageant parfois entre plusieurs communes, ils exercent un rôle essentiel, comme beaucoup d’entre nous pourront certainement en attester au regard de leur expérience d’élus locaux.

si elles ne le sont pas déjà. Ces problèmes se traduisent en particulier par une pyramide des âges vieillissante annonçant d’importants départs à la retraite, qui devront être anticipés si nous voulons éviter l’émergence de nombreuses fragilités dans l’administration communale de demain. Par ailleurs, la profession de secrétaire de mairie requiert une forte polyvalence et une technicité administrative bien plus grande que par le passé. Pourtant, malgré la nature changeante du travail effectué, plus de 60 % des secrétaires de mairie appartiennent toujours à la catégorie C et plus de 20 % à la catégorie B. Aux quatre cadres d’emploi concernés par cette répartition s’ajoute une forte part de contractuels. Le résultat est une dispersion des statuts et des situations, ainsi qu’une inadéquation entre le niveau de responsabilité réel

Le texte que nous avons voté prévoyait en particulier de faciliter la promotion interne, mais aussi de permettre de recruter des contractuels dans les communes de moins de 2 000 habitants, contre 1 000 aujourd’hui, ou encore de mettre en place un cadre plus rigoureux de formation des secrétaires de mairie. Enfin, il a été décidé d’inscrire la fonction dans le code général des collectivités territoriales, en mettant en particulier en avant le titre de « secrétaire général de mairie », permettant de reconnaître à sa juste valeur l’importance de la fonction et de la distinguer de ce qui relève du seul secrétariat du maire. Nous constatons avec satisfaction que les députés ont largement partagé notre appréciation de la question, retenant des dispositifs proposés par le Sénat, sans divergences fondamentales, avant d’unanimement voter le texte.

Un autre sujet concernait les facilités données de la promotion des agents. Avec le rétablissement de l’article 2 , nous avons obtenu le maintien d’un mécanisme favorisant également la promotion interne des agents des catégories B vers la catégorie A,

En effet, les secrétaires de mairie sont les piliers de notre administration locale. Leur rôle est essentiel : gardiens des procédures administratives, agents de première ligne, accueillant nos concitoyens avec professionnalisme et empathie. Nos secrétaires de mairie incarnent l’esprit du service public, bien souvent dans l’ombre, mais avec une influence considérable sur le bon fonctionnement de nos C’est pourquoi il était impératif de reconnaître leur importance en créant une attractivité réelle pour ce métier où les difficultés de recrutement sont réelles, avec plus 1 900 postes vacants. Nous soulignons les avancées : création d’une voie de promotion interne obligatoire, création d’une formation initiale qualifiante, bénéfice d’un avantage spécifique d’ancienneté, facilitation de la promotion interne. Les maires de ces communes nous font quotidiennement part de leur difficulté. Je tiens ici à rappeler que les élus de ces petites communes sont souvent le catalyseur de la cohésion sociale et restent les acteurs indispensables à la vitalité de nos territoires, loin de la vision souvent mondialisée du Gouvernement. Les communes rurales sont le cœur battant de nos traditions et de notre patrimoine. Vous les avez trop souvent oubliés ces dernières années, en leur laissant le sentiment d’être souvent bien seuls face aux difficultés de leurs administrés, portant votre attention et les ressources sur les grands centres urbains. Pour une fois, monsieur le ministre, vous semblez avoir entendu et écouté l’importance du rôle de secrétaire de mairie dans le quotidien d’un maire et d’une municipalité rurale.

Nous sommes attachés au pragmatisme et nous voterons toujours ce qui peut améliorer le quotidien de nos compatriotes. Nos collègues à l’Assemblée nationale ont défendu et adopté cette avancée, notamment le député Pierrick Berteloot, fortement engagé sur cette question. Dans cette continuité, nous voterons également en faveur de cette proposition de loi. Notre boussole sera toujours l’intérêt du peuple de France.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous remercions les rapporteurs de la commission des lois et l’ensemble des parlementaires qui ont participé à l’élaboration de ce texte commun.

La commission mixte paritaire est parvenue à un accord sur les dispositions du texte restant en discussion. Nous nous en réjouissons. Il est important de valoriser le métier de secrétaire de mairie. Essentiels à la vie de nos communes,

de budget. Secrétaire de mairie est également un métier sensible, qui implique de bâtir une relation de confiance avec les élus. C’est d’autant plus vrai dans les très petites communes, où le maire est parfois le seul interlocuteur donc urgent de proposer des mesures concrètes pour revaloriser ce métier et renforcer son attractivité. Cela a été rappelé, un tiers des secrétaires de mairie partiront à la retraite au cours des huit prochaines années. Notre boussole au cours de l’examen de ce texte a été d’introduire de la souplesse dans les processus d’embauche, de sécuriser le parcours des secrétaires de mairie et de leur permettre de progresser en termes de statut et de salaire. Ce texte est un premier pas satisfaisant. Nous devons continuer dans ce sens, afin d’endiguer la pénurie de secrétaires de mairie qui s’annonce et de valoriser ces agents à la hauteur de l’importance de leurs missions. Le groupe Les Indépendants – République et Territoires soutient l’adoption de ce texte. Conformément

Merci